La séance est ouverte.

au moins une réponse positive parmi les voeux qu'ils ont formulés. formulés. Nous partageons votre objectif d'une obtention par les deux tiers des jeunes d'un voeu d'admission avant le début des épreuves du baccalauréat. Le groupe La République En Marche tient à féliciter les équipes du ministère, que les équipes pédagogiques, qui ont dû s'approprier en un temps record ce nouvel outil et analyser les situations. Elles méritent notre respect, car de leur engagement dépend la réussite des étudiants.

Nous ne regrettons pas le système précédent, qui était une impasse. Et celles et ceux qui avaient accepté comme outil le tirage au sort ne sont pas les mieux placés pour donner des leçons

Les réseaux sociaux se sont fait l'écho de situations, parfois difficiles à déchiffrer, pour les jeunes et leurs familles. Il vous reste dix secondes, pas d'amplifier les faux messages, parfois complaisamment relayés, mais les inquiétudes sont légitimes. Madame la ministre,

font leur choix, parce que nous avons voulu leur donner le choix, d'autres lycéens reçoivent des propositions et peuvent à leur tour choisir. La dynamique fonctionne, et Parcoursup

de réussite en licence. Ce n'est pas l'ambition de ce gouvernement. Nous souhaitons que les jeunes non seulement accèdent à l'enseignement supérieur, mais surtout qu'ils y réussissent, car nous avons besoin d'une jeunesse formée et diplômée. La parole

vous avez récemment accepté que Total exploite sur le site de La Mède quelque 300 000 tonnes d'huile de palme brute, pour une production annuelle de 500 000 tonnes de biocarburant. biocarburant. Or cette situation peut être très lourde de conséquences. En effet, elle pourrait priver les producteurs français d'oléagineux d'un débouché durable, qui a permis de bâtir une filière performante, assurant à la fois sa vocation de nourricière principale de l'agriculture et sa participation à la transition énergétique. L'utilisation d'huile de palme importée suscite de lourdes inquiétudes sur le plan tant agricole qu'écologique. D'une part, cela pourrait concurrencer, voire déstabiliser, les filières nationales bâties autour des productions biodiesel de colza et de tournesol, qui valorisent les productions de proximité. D'autre part, la culture de l'huile de palme est la principale cause de déforestation en Asie du Sud-Est. Cette décision semble en parfaite contradiction avec l'axe 15 de votre plan Climat, visant à lutter contre la déforestation importée. L'impact immédiat de cette production sur la filière de colza peut être considérable, en entraînant une perte de 400 000 hectares, soit une diminution de 27 % des surfaces actuelles. La filière biocarburants européenne et française constitue une source de protéines qui nous permet d'être moins dépendants du soja américain, très majoritairement OGM. À l'heure où il est question de défendre l'agriculture française, pour mieux lui permettre de répondre à des défis décisifs, cette annonce semble en contradiction avec l'ambition portée par le Gouvernement. Monsieur le ministre d'État, la filière française de biocarburants est essentielle pour notre agriculture.

un accord a été conclu entre Total et le gouvernement précédent pour transformer cette raffinerie en bioraffinerie, afin de préserver 450 emplois. Total a effectué plusieurs centaines de millions d'euros de travaux.

à 300 000 tonnes la consommation annuelle d'huile de palme, pour encourager plutôt la hausse, d'année en année, de l'utilisation des huiles usagées. Le plus important, parce que c'est le sens de l'histoire- nous y travaillons au niveau européen -, c'est de faire en sorte que l'Europe

Avec un slogan qui sonne comme une publicité pour la Française des jeux, « une chance pour chacun », le Président de la République a enterré le rapport Borloo. Mais la chance n'a rien à voir là-dedans Dans mon département de Seine-Saint-Denis, un rapport parlementaire pointe que les taux de chômage, de pauvreté et de difficultés scolaires sont bien supérieurs aux moyennes nationales. On compte ainsi deux fois moins de magistrats au tribunal d'instance d'Aubervilliers que dans un tribunal parisien équivalent. Autre exemple, le moins bien doté des établissements scolaires parisiens est mieux loti que le plus doté des établissements de la Seine-Saint-Denis. Contrairement aux idées reçues,

Sans parler de l'accès à la santé, au logement ou à l'emploi ... Bref, tous les sas d'entrée dans la République sont défaillants. La banlieue et ses habitants sont souvent discriminés et stigmatisés. Ils sont maintenant méprisés. Pis, ils sont mis au ban de la République, car c'est toute la promesse d'égalité que vous avez enterrée. Nous avons été abasourdis par les propos du Président de la République, lorsqu'il a parlé de « deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers Au-delà du mépris pour Jean-Louis Borloo, c'est nier que le rapport est issu d'une concertation avec des centaines d'élus de tous bords politiques, notamment ceux qui ont participé à l'appel de Grigny, des associations et des citoyens. que leur espoir, que vous avez enterré hier, c'est leur travail que vous avez nié sur le terrain. Votre politique, c'est à chaque coup un ticket gagnant pour les nantis de ce pays. Pour les autres,

! Vous avez parlé de l'enterrement du plan Borloo. Non ! Jean-Louis Borloo lui-même s'est dit satisfait des orientations du Président de la République. en avoir suivi l'élaboration, avec les groupes de travail que nous avons mis en place, je puis vous dire que

Les fonctionnaires, ces sentinelles de la République, consacrent leur vie à la défense du service public et ne comptent pas leurs heures pour garantir la cohésion sociale. La fonction publique incarne des valeurs auxquelles nos concitoyens sont viscéralement attachés : la laïcité, l'égalité, la gratuité, l'indépendance, la solidarité. Ne gâchons pas cette richesse humaine ! Contrairement à ce que laissent entendre vos, les fonctionnaires ont fait beaucoup d'efforts et ont subi patiemment le gel du point d'indice. Malgré cela, vous bloquez toute revalorisation, pourtant prévue par la précédente majorité. Vous ne choisissez la modernisation du service public que sous l'angle strictement budgétaire, alors que l'efficacité et la qualité d'un service public s'évaluent d'abord socialement, pour la simple et bonne raison qu'il est notre bien commun, notre, qui dépasse les totems de la performance et de la rentabilité. Entendez-le, monsieur le secrétaire d'État, cette idée du service public demeure une idée d'avenir, profondément moderne. Entendez les organisations syndicales, qui vous demandent à l'unisson de sortir du raisonnement comptable à sens unique. La fonction publique n'est pas un bloc monolithique. Elle a démontré sa capacité à réformer ses pratiques. Mais, au lieu d'augmenter ce patrimoine de tous que représentent nos services publics, vous enrichissez les plus nantis. Vous avez récemment reculé sur la remise en cause frontale du statut. Mais qu'en sera-t-il dans quelques semaines, après la publication du rapport du Comité Action publique 2022 ? Vous affichez l'ambition de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Quelle est la plus-value de cette réforme pour notre pays, qui attend de connaître les secteurs concernés ? Y aura-t-il moins de personnels dans les hôpitaux, dans les EHPAD, moins d'agents de police, moins de professeurs, moins d'agents territoriaux ? territoriaux ? Ma question est simple : avez-vous des propositions concrètes à formuler pour enrayer cette logique destructrice, repenser la modernité du service public et lui redonner un véritable avenir ?

bien volontiers à l'hommage appuyé que vous venez de rendre à nos fonctionnaires, quelle que soit la fonction publique dans laquelle ils exercent. Vous le savez, le Gouvernement a lancé à l'automne dernier le programme Action publique 2022, auquel nous avons assigné un objectif : adapter l'action publique, pour qu'elle permette de rendre un meilleur service à nos usagers et qu'elle puisse répondre avec la plus grande efficacité aux défis du XXI siècle. Nous suivons une méthode, celle de la discussion avec l'ensemble des organisations syndicales, selon un calendrier d'une année. De très nombreux chantiers ont été ouverts par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt : rémunération au mérite, extension du domaine des contrats, formation et plans de départ volontaire, réforme des instances de représentation. D'autres réflexions, d'ailleurs issues de demandes des organisations syndicales elles-mêmes, viennent enrichir le débat, en particulier la question sensible de l'attractivité des concours. Nous avons, vous le savez également, un agenda. À la demande des organisations syndicales, le rendez-vous, initialement prévu au mois d'octobre prochain, a été avancé au mois de juin. Pour ce qui concerne le pouvoir d'achat, je rappelle que le gel du point d'indice ne date pas de ce quinquennat et qu'une augmentation du point

les attaques reprennent, entraînant la mort d'animaux et la baisse de la lactation, due au stress. Les éleveurs sont de plus en plus enclins à garder leurs animaux à l'intérieur des bergeries. Alors que nous sommes classés au patrimoine mondial de l'UNESCO pour l'agropastoralisme, le loup perturbe ce fragile équilibre. En effet, sans brebis, point de biodiversité. Le commissaire européen s'est empêtré dans des propositions technocratiques, et il a même laissé penser que chaque État avait la latitude nécessaire pour gérer ses populations de loups Face au désarroi de nos éleveurs, nous ne comprenons pas les contradictions entre la directive Habitats-faune-flore et la convention de Berne. Monsieur le ministre d'État, au vu de la dont l'espèce n'est plus menacée, et de la biodiversité, dont nous savons tous qu'elle est en danger sur notre planète, quelles mesures comptez-vous prendre pour protéger l'agropastoralisme ?

il y a des dossiers particulièrement difficiles à porter ... Entre Brigitte Bardot qui m'invective toutes les semaines parce qu'elle voudrait que l'on ne touchât pas à un seul loup et quelques éleveurs- pas tous ! -qui me vouent aux gémonies et aimeraient que l'on éradique l'ensemble des loups, vous comprendrez que le compromis est compliqué. Il en va du respect de la biodiversité naturelle comme du respect de la diversité culturelle : on ne peut avoir d'affection sélective.

un changement de méthode- une philosophie de mobilisation générale envers les habitants des quartiers prioritaires se traduisant par une série de mesures. Je n'en cite que quelques-unes : 15 000 places de stage pour les collégiens de la classe de troisième, la création de 30 000 places de crèche pour faciliter le travail des femmes,

C'est un camouflet et une déception sévère et amère pour les élus locaux, pour les associations de proximité, mais aussi pour les habitants, auxquels on doit redonner de l'espoir et l'envie de la France. Pour tous ceux-là, monsieur le ministre, il faut avant tout rétablir l'ordre et la sécurité, de manière totale et pérenne, en luttant contre l'économie souterraine et les trafics qui gangrènent le tissu social, en mettant fin aux actes barbares des voyous, au communautarisme, au prosélytisme islamique

La parole est à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la cohésion des territoires.

son propos par la question de la sécurité, en rappelant que l'engagement de ce gouvernement était d'augmenter de 1 300 postes l'effectif des fonctionnaires de police

Mardi dernier, nous apprenions que le Président de la République, s'inspirant, sans pour autant le reprendre à son compte, du rapport Borloo sur les banlieues, dévoilait une série de mesures visant à aider les quartiers défavorisés. Les propositions de Jean-Louis Borloo ont été très bien accueillies par les élus locaux. Les médias, également, ne s'y sont pas trompés et leur ont réservé, à juste raison, un très large écho. Dans le même temps, nos territoires ruraux souffrent pareillement des mêmes maux- pauvreté, chômage, violence, recul des services publics de proximité -, mais ne semblent pas du tout constituer une priorité pour le Gouvernement. Il conviendrait pourtant d'entendre cette souffrance qui monte de nos campagnes. Elles aussi manquent cruellement de moyens depuis un moment déjà. La France, mes chers collègues- c'est une phrase que je prononce dans cette enceinte avec force, car je sais qu'elle y sera entendue -ne se réduit pas aux seules grandes métropoles. Notre pays est une mosaïque de territoires qui racontent notre histoire et dont les habitants méritent également toute l'attention de la Nation. La Haute Assemblée, tendances confondues, est résolument et tout entière à leurs côtés. Elle l'a montré tant de fois sur tant de sujets. Aussi, monsieur le ministre, qu'attendez-vous pour mettre en place une politique ambitieuse en faveur des territoires ruraux ? À quand un grand plan Ruralité ?

Voilà quelle est la réalité. C'est vrai ! Ce dont nous avons besoin, ici et ailleurs, c'est de déterminer un certain nombre d'actions pour améliorer la situation des territoires ruraux qui sont en décrochage. Il y en a, j'en connais et je suis bien placé pour le savoir. Le travail réalisé par le Gouvernement sur le numérique par exemple, qui est en train de porter ses fruits et qui est important et même indispensable pour l'avenir de ces territoires, constitue un plus. Le travail que nous menons sur les internats d'excellence, celui que nous accomplissons sur la loi concernant l'agriculture, tout cela est important ! Dire que rien ne se fait et que nous n'aurions aucune vision n'est pas vrai. De grâce, arrêtons ces clichés ! Que nous ayons des sensibilités différentes, une approche différente, peut-être

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question concerne nos concitoyens en situation de handicap, en lien avec l'examen prochain de la proposition de loi du député Philippe Berta relative à l'amélioration de la prestation de compensation. Il est vrai que, depuis la loi de 2005, le droit à compensation a peu progressé, même si l'on doit souligner la revalorisation récente de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH. Les personnes en situation de handicap et leurs familles avaient pourtant fondé de grands espoirs sur cette loi. Elles sont aujourd'hui très inquiètes.

au-delà de l'impact très négatif de la diminution du nombre de contrats aidés sur l'action des auxiliaires de vie scolaire, les AVS, j'ai été interpellé sur les difficultés rencontrées par les personnes souffrant de troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Ces troubles ne sont pas toujours assimilés à un handicap, ce qui peut conduire à un refus d'obtention d'aménagement des modalités de passation des examens et concours, qui plus est dans un contexte où la réglementation laisse place à des interprétations divergentes selon les rectorats ou les ministères de tutelle porte enfin sur les conditions de vie, car, si l'on peut se féliciter de la suppression à venir de la barrière des soixante-quinze ans, l'on ne peut que regretter la timidité de la proposition de loi concernant la question sensible du reste à charge, inscrite dans la loi de 2005, mais restée lettre morte depuis Si ces problématiques ne sont pas récentes, il n'en reste pas moins que certaines décisions prises par le gouvernement actuel fragilisent des personnes handicapées dans un contexte où leurs associations questionnent la méthode de concertation du Gouvernement. Je vous renvoie sur ce point à la tribune publiée dans du 5 mai dernier. Aussi, j'aimerais connaître quelles mesures opérationnelles le Gouvernement entend prendre pour remédier à ces difficultés et enfin mettre en application ce qui a été annoncé comme une priorité par M. le Président de la République. La parole

vous l'avez dit, le Président de la République a souhaité faire de l'inclusion des personnes en situation de handicap une priorité d'action. Il l'a fait avec une double conviction : celle qu'il y avait encore beaucoup à accomplir pour faire pleinement la place aux différences et celle que se jouaient dans la question de l'intégration des plus fragiles un changement de notre regard et un véritable enjeu de société, au bénéfice du plus grand nombre. Animée de cette ambition très forte, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, met en oeuvre depuis un an cette politique transversale, notamment est rattachée à M. le Premier ministre pour être plus opérationnelle et plus efficace. Le mode opératoire est commun à l'ensemble du Gouvernement : entrer dans une culture de résultats et d'efficacité. Les résultats de la première année sont nombreux : renforcement de l'accompagnement des élèves en situation de handicap, avec la sanctuarisation de 50 000 contrats aidés dans l'éducation nationale ; création de 8 000 emplois pérennes à la rentrée dernière ; revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés, pour atteindre 900 euros dès 2019 déploiement du dispositif de l'emploi accompagné dans l'ensemble des régions ; mise en place d'un guichet unique ; généralisation de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » à l'ensemble des régions pour garantir une réponse aux fragiles. Bien sûr, ces avancées ne permettent pas de répondre à toutes les difficultés, qui sont parfois anciennes. Le Gouvernement s'est donc engagé dans de véritables actions de transformations structurelles, en particulier avec les chantiers de l'école inclusive et de l'entreprise inclusive. Nous aurons l'occasion de rediscuter

professionnel. Les concertations pour construire ces projets se font avec les personnes en situation de handicap et leurs représentants, en particulier le Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, les élus et les habitants des quartiers attendaient un engagement majeur du Président de la République en faveur des banlieues. Quelle déception ! Aucune proposition significative du rapport Borloo n'est reprise, et rien n'est proposé à la place. Emmanuel Macron ne veut pas écouter, il ne veut pas voir la réalité en face. D'un côté, il sous-estime la gravité de la situation dans certains quartiers- plusieurs centaines conséquent, il n'engage ni stratégie opérationnelle ni moyens financiers et humains pour résoudre les problèmes. De l'autre, il refuse de reconnaître les réussites- il y en a ! en a ! -, pour mieux disqualifier la politique de la ville et justifier les coupes budgétaires qui pénaliseront les catégories populaires et les quartiers. Il y en a déjà : la baisse des APL, les ponctions massives sur le logement social, la suppression des contrats aidés et même la suppression de la délégation à la mixité à la mixité sociale. Le miracle viendrait du retour au droit commun. Toutefois, celui-ci n'a jamais été abrogé, et s'il est nécessaire, il n'est pas suffisant. La simple mise en oeuvre de la sécurité au quotidien, à des échéances bien éloignées, ne suffira pas à rétablir une vie normale là où la situation est très dégradée. Il faut des moyens pour la justice, la prévention, et une mobilisation générale. Le seul dédoublement en CP et CE1 ne suffira pas à la réussite du cursus scolaire de ces enfants. Il faut des moyens supplémentaires. Sans des ressources nouvelles pour l'éducation populaire et la vie associative, nous n'arrêterons pas les dérives qui, trop souvent, éloignent certains quartiers de notre République. Oui, c'est bien un rattrapage et une reconquête républicaine qui s'imposent. C'est bien une nouvelle étape de la politique de la ville qu'il faut ouvrir, et non son enterrement. Le Président de la République a manqué le rendez-vous, nous ne pouvons en rester là ! Monsieur le ministre, quelles actions concrètes le Gouvernement compte-t-il prendre pour les banlieues ?

annoncée au plus haut niveau. Voilà quelle est la réalité ! On peut toujours dire que ce n'est pas assez et qu'il n'y a pas assez d'argent. Mais quel est le résultat ? Ce n'est pas cela qui a changé la situation. Je vous demande donc simplement un peu de sérénité et d'engagement, parce que nous avons besoin d'être rassemblés face au danger communautariste. Voilà quelle est la réalité

d'abord, le non-respect des valeurs limites de pollution atmosphérique, et ensuite, un manquement à l'obligation de prendre des mesures pour limiter ces dépassements. Visiblement, le plan que vous avez adressé à la Commission européenne le 13 février dernier n'a pas convaincu. C'est un nouvel et très sérieux avertissement, après la décision du Conseil d'État de juillet 2017, qui vous exhortait à agir. Ma question est simple, monsieur le ministre d'État : puisque l'heure est à l'action, quelles mesures envisagez-vous de prendre pour répondre à cet enjeu de santé publique, qui est, avec le réchauffement climatique, la préoccupation environnementale prioritaire

années d'aménagement du territoire et de politique de transport qui n'ont pas fait de cette question une priorité, sauf à fermer demain matin certaines activités industrielles, interdire certains modes de chauffage et retirer des millions de véhicules de la circulation, je ne sais pas le faire Je vous le dis très franchement, je ne sais pas le faire dans un temps court. Ce n'est pas pour autant que nous baissons les bras. Je pars d'une situation critique, qui n'est ni acceptable ni tolérable, parce que, vous l'avez rappelé, cela touche à la santé, et toujours à celle des plus vulnérables.

diesel. Je suis désolé de vous le dire, mais les particules fines font partie des sujets de santé publique ! La prime à la conversion a d'ores et déjà permis à 45 000 véhicules polluants d'être remplacés

dont le niveau est aujourd'hui trop élevé, plutôt que de faire de la « com » les jours de pic de pollution. Stigmatiser le seul automobiliste pour se donner bonne conscience ne constitue pas une politique à la hauteur de l'enjeu. L'État a en effet une responsabilité éminente au regard des politiques de santé publique et de préservation de l'environnement. Il ne peut pas et ne doit pas se dérober. Il doit enfin élaborer une politique concertée avec les quatre grandes familles d'émetteurs que sont l'habitat et le résidentiel, l'agriculture, les transports et l'industrie. J'entends que l'État ne peut pas tout, mais il a aussi pour mission d'accompagner les territoires et les collectivités territoriales, au travers des plans de protection de l'atmosphère et des plans climat-air-énergie territoriaux. Il peut aussi se nourrir des travaux des assemblées parlementaires,

À l'occasion de votre premier budget, vous avez choisi de privilégier l'écologie punitive, en augmentant systématiquement les taxes dites « comportementales ». Il faut conclure ! Aujourd'hui, relevons ce beau défi, celui de l'écologie positive, qui fait appel à l'intelligence collective

ont été rejetés, au motif qu'un groupe de travail serait mis en place en vue de revoir ce dispositif pour 2019. Depuis lors, j'ai sollicité votre ministère, ainsi que celui de la cohésion des territoires et celui des comptes publics et, malgré toute votre écoute, je n'ai pas eu, à ce jour,

ce territoire en difficulté est devenu contributeur net au Fonds et reverse donc plus à l'État qu'il n'en reçoit de dotations. Il est ainsi ponctionné par ce fonds dit « de péréquation » à hauteur de pratiquement 50 % de ses ressources fiscales intercommunales. Madame la ministre, vous qui connaissez parfaitement les collectivités locales et les réalités des territoires, vous devez corriger cette injustice fiscale ! Dans l'attente d'une réforme structurelle du FPIC,

Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie et des finances. Le ministère des affaires étrangères et du développement international a mis 285 agents à la disposition du réseau des alliances françaises à l'étranger, pour une masse salariale d'environ 30 millions d'euros. Il s'agit de 211 expatriés, directeurs et chargés de mission, soit 18 % des effectifs globaux du réseau culturel extérieur de la France.

à l'étranger ; les frais de scolarité ont augmenté, et les enfants à besoins éducatifs particuliers ne seront toujours pas pris en charge. M. Bruno Le Maire a annoncé dimanche dernier sur une chaîne télévisée qu'il souhaitait que la taxe d'habitation soit maintenue sur les résidences secondaires ; cela concerne beaucoup de Français de l'étranger,

de l'enseignement français à l'étranger ou des alliances françaises, nous avons exprimé une volonté forte. Le Président de la République a pris des engagements très clairs lors de son discours à la communauté française de Tunis, en février dernier.

l'apprentissage du français et le rayonnement de la France au travers de la culture et de l'innovation. De ce point de vue, les crédits alloués sont également au rendez-vous, puisque, en 2018, 35 millions d'euros sont consacrés aux alliances françaises, ce qui est exactement en ligne avec ce qui leur était destiné précédemment.

un très grand serviteur de l'État, nous allons pouvoir progresser pour faire en sorte que les alliances françaises soient mieux représentées dans la structure de tête, et pour rapprocher ces dernières de l'Institut français, selon des modalités qui restent

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le Premier ministre.

Le communautarisme ne cesse d'étendre son emprise, que ce soit à l'université, à l'école, dans les quartiers, mais aussi dorénavant dans les syndicats, les entreprises et, hélas, les services publics. La France, ce n'est ni le communautarisme ni le multiculturalisme. Ne nous y trompons pas : la visibilité de certains signes religieux constitue un message à valeur politique, celui du refus de l'intégration dans notre République et du rejet de ses valeurs émancipatrices de liberté, d'égalité, de fraternité, mais également de laïcité. Les « accommodements raisonnables », voire électoraux, qui semblent satisfaire certains, ou le « machisme » que semblent voir d'autres, c'est le recul de la République et du droit des femmes. Au Sénat, nous avons choisi de mener le combat : propositions de loi pour renforcer la laïcité à l'école et à l'université, ou encore amendements au projet de loi sur les violences faites aux femmes. Le Sénat sera toujours fort pour défendre la République ; le Sénat sera toujours le dernier rempart des valeurs de la France. Ma question est donc simple. Quelle société le Gouvernement veut-il vraiment ? Va-t-il accepter encore longtemps la part croissante des emprises communautaires de tous types dans notre pays, si contraires à nos valeurs et à notre pacte national, ou entend-il agir avec fermeté pour lutter contre ces régressions ?

qui a conçu la laïcité française comme une laïcité de liberté : certes, l'État ne reconnaît aucune religion, mais chaque citoyen doit aussi pouvoir exercer son culte dans de bonnes conditions, ou encore n'en exercer aucun. ans après l'entrée en vigueur de cette loi, le Gouvernement est plus que jamais décidé à en appliquer les principes ; rien que la loi de 1905, toute la loi de 1905. Le communautarisme, quant à lui, doit être combattu avec fermeté, car il n'existe dans notre pays qu'une seule communauté, celle de la République française,

quartiers et partout où nous devons le faire. Nulle part, nous ne pouvons accepter que des préceptes religieux veuillent l'emporter sur les lois de la République. Nulle part, nous ne pouvons nous résigner à ce que la République ne donne pas aussi sa chance à chacun. Nous serons sur tous les fronts, monsieur le sénateur, la sécurité, l'emploi, l'éducation. Nous agissons pour améliorer le quotidien et l'avenir de nos concitoyens, dans le respect de la laïcité.

Une France forte dans ses valeurs n'a pas peur d'intégrer. Nous voulons une France ouverte dans l'Europe, mais unie dans ses principes et dans ses valeurs, sur tout le territoire que, le mercredi 30 mai prochain, nous pourrions reporter l'ouverture de la séance à seize heures, afin de permettre à la commission des affaires sociales d'examiner, dans le cadre de la législation en commission, la proposition de loi relative à l'autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées. Par ailleurs, le délai limite de dépôt des amendements sur la proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extraparlementaires et à simplifier les modalités de leur nomination, également examinée selon la procédure de législation en commission, pourrait être repoussé au mardi 5 juin 2018,